La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mardi 30 avril 2024 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n’y a pas d’observation ?… Le procès verbal est adopté. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions orales. La parole est à M. Stéphane Sautarel, la santé et des solidarités. Monsieur le ministre, comme vous le savez, les praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue) qui veulent exercer en France doivent passer par une lourde et longue procédure administrative avant de pouvoir pratiquer librement leur profession épreuves de vérification des connaissances (EVC), parcours de consolidation des compétences (PCC) – celui ci nécessite d’effectuer deux ans de fonctions hospitalières en qualité de praticien associé –, puis demande d’autorisation d’exercice de la profession en France. C’est seulement à l’issue de ce long processus administratif et pratique que les médecins étrangers peuvent exercer librement dans Le Président de la République s’est engagé le 16 janvier dernier à sécuriser la situation des Padhue. Celle des candidats non lauréats fait encore l’objet de décisions dérogatoires et temporaires et fait suite à la fin d’un régime dérogatoire qui existait jusqu’au 31 décembre 2023. Cependant, la situation de ces médecins étrangers ne peut plus faire l’objet de régimes dérogatoires successifs : il faut des mesures efficaces et définitives. Dans le Cantal, alors que nous manquons cruellement de médecins et que nous sommes confrontés à des déserts médicaux, comme bien d’autres territoires ruraux, des médecins ou des dentistes étrangers candidats à l’installation rencontrent des difficultés pour exercer et en sont souvent empêchés. est pourtant une véritable solution d’urgence pour pallier ou tenter de pallier le manque de médecins. Cela permettrait de rendre un véritable service à nos populations, qui ont droit, comme tous les Français, à un accès aux soins. Monsieur le ministre, que comptez vous faire pour assouplir et faciliter le travail des médecins étrangers à diplôme hors Union européenne, ainsi que pour accélérer et simplifier leur installation ? La parole

Monsieur le sénateur Stéphane Sautarel, l’autorisation d’exercice pour les praticiens à diplôme hors Union européenne est à la fois un enjeu individuel pour les intéressés et une mesure permettant

Il n’existe qu’une seule voie d’accès permettant l’obtention du plein exercice : les praticiens à diplôme hors Union européenne doivent se présenter présenter aux épreuves de vérification des connaissances et, à leur issue, réaliser un parcours de consolidation des compétences de deux ans. Ce concours a lieu chaque année. Une refonte de la procédure concernant les Padhue est actuellement engagée, afin de fluidifier leur parcours de demande d’autorisation d’exercice. Depuis la loi du 27 décembre dernier, les praticiens peuvent disposer d’une autorisation temporaire d’exercice de treize mois en attendant de passer le concours, et celle ci est renouvelable une fois en cas d’échec. Par ailleurs, les praticiens qui exerçaient déjà en France au moment des résultats du concours de 2023 ont pu bénéficier d’une affectation prioritaire sur leur établissement employeur. D’autres évolutions seront mises en œuvre à compter de la saison 2024. les épreuves de vérification des connaissances qui auront lieu à l’automne permettront notamment de prendre en compte l’expérience acquise sur le territoire français par ces praticiens. Par ailleurs, en application de l’article 36 de la loi du 27 décembre 2023, la durée et le parcours de consolidation des compétences seront aménagés. Le praticien lauréat du concours pourra se voir délivrer une autorisation de plein exercice à la suite d’un stage d’évaluation, après l’examen de son dossier par une commission d’autorisation d’exercice. Par toutes ces mesures, j’ai la conviction que nous facilitons la régulation et la régularisation des praticiens à diplôme hors Union européenne tout en veillant à la qualité de leurs compétences, gage de la qualité des soins.

de la santé et des solidarités étaient suspendues, dans l’attente de la finalisation des arbitrages par le cabinet du Premier ministre. Cette décision affecte directement le remboursement du dispositif « cantine à 1 euro ». Cette mesure de tarification sociale mise en place par l’État en avril 2019, à destination des communes rurales de moins de 10 000 habitants, permet aux enfants des familles modestes de déjeuner dans les cantines scolaires pour 1 euro maximum. Depuis le mois de février dernier, le ministère n’a pu abonder la trésorerie du dispositif. Les demandes de remboursement sont donc suspendues, en attendant d’être traitées par l’Agence de services et de paiement (ASP), qui gère ce dispositif.

Il avait été précisé aux élus locaux que le principe de remboursement ne serait pas remis en cause. Compte tenu de cet important retard et de l’absence totale d’informations régulières délivrées sur l’évolution de la situation, les élus sont en droit de craindre le pire, à savoir que cette suspension de paiement ne soit le prélude à une suppression du dispositif. Monsieur le ministre, êtes vous en mesure de nous indiquer quand les arbitrages attendus seront rendus, et si ce dispositif reprendra son fonctionnement normal dans la foulée ? La parole est à M. le ministre

Pour preuve, en 2023, ce sont près de 2 500 communes ou regroupements de communes qui ont reçu une subvention de 3 euros par repas, servi à un tarif social de 1 euro ou moins. Autre chiffre significatif, plus de 15 millions de repas servis à tarif social ont été subventionnés par l’État et, en moyenne, quelque 194 000 élèves ont pu rester ou retourner à la cantine grâce au dispositif sur l’année scolaire 2022 2023. Comme votre question le souligne, une évolution supplémentaire vient enrichir la mesure depuis janvier 2024, avec le versement d’une subvention qui peut passer de 3 à 4 euros par repas – c’est « le bonus Égalim lorsque la collectivité s’engage à tout mettre en œuvre pour atteindre l’objectif de la loi Égalim visant à introduire dans les cantines 50 % de denrées locales et de qualité, dont 20 % de bio. Cette bonification peut être demandée dès maintenant par les communes qui bénéficient d’ores et déjà du dispositif ou par

Élisabeth Borne et, à ce titre, est confortée jusqu’en 2027. L’Agence de services et de paiement gère ce dispositif pour le compte de l’État. C’est avec cette agence que les communes passent la convention pluriannuelle et que les services de l’État ont préparé ont préparé la prolongation et l’évolution de la mesure, pour être en ordre de marche dès janvier 2024. Il est confirmé, tout d’abord, que les collectivités qui ont déjà passé une convention pluriannuelle peuvent la renouveler auprès de l’Agence de services et de paiement au moment de son échéance, sous réserve de continuer à respecter les critères d’éligibilité, et, ensuite, que les collectivités le souhaitant peuvent signer à tout moment un avenant à la convention en cours pour bénéficier du bonus Égalim, sous réserve d’avoir pris connaissance des engagements qui y sont associés. Toutes ces informations et les modèles d’avenant

Je suis bien conscient que les erreurs de calcul du Gouvernement concernant les dépenses publiques le conduisent aujourd’hui à trouver des économies dans la panique… Je vous mets néanmoins en garde contre la tentation de mettre une fois de plus en difficulté les collectivités locales et nos concitoyens ! La tarification sociale des cantines est une mesure juste, à laquelle de nombreuses communes rurales ont recours, et elle est destinée à bénéficier aux enfants des familles modestes. Les priver d’un tel dispositif serait aller à l’encontre de la justice sociale. Si l’État a besoin d’argent, s’il connaît des difficultés de trésorerie,

et de la prévention. Monsieur le ministre, les dérives commerciales récentes d’un certain nombre de centres de santé dentaires ont eu de graves conséquences, tant sur la qualité et la sécurité des soins bucco dentaires que sur leur coût pour l’assurance maladie. Parmi elles, je citerai des cas de mutilation et la réalisation d’actes non nécessaires et même, parfois, fictifs. Le Parlement a adopté la loi du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. pour que ce texte soit pleinement efficace, encore faut il que les six mesures réglementaires qui l’accompagnent soient appliquées rapidement… Or, à ce jour, elles n’ont pas été mises en œuvre. La loi votée l’année dernière accroît les missions de contrôle des agences régionales de santé (ARS), avec notamment le rétablissement de la procédure d’agrément préalable des centres. Cette procédure avait été supprimée, faute de moyens suffisants pour les ARS, par la loi portant du 21 juillet 2009. Cette suppression a sans aucun doute favorisé les dérives constatées ces dernières années, dénoncées par les professionnels de santé chirurgiens dentistes. Il convient donc de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de traduire l’esprit de la loi en actes. Afin de m’assurer que le texte voté l’année dernière ne soit pas privé d’effets, je souhaite savoir, monsieur le ministre, à quelle échéance seront publiées les mesures réglementaires d’application et quels sont les moyens financiers et humains qui ont été alloués aux ARS pour conduire les opérations qui leur ont été confiées par le législateur sur les centres de santé. La parole est à M. le ministre

dans certains centres – vous avez cité les centres dentaires, mais on pourrait évoquer également les centres d’ophtalmologie. Ces dérives portent atteinte à la solidarité nationale, comme vous l’avez rappelé. Vous avez pu constater que nous avons d’ores et déjà agi. L’assurance maladie a ainsi décidé

sont accompagnées, sur les plans méthodologique et juridique, par les services du ministère, ce qui permettra aux ARS d’appréhender au mieux le traitement des dossiers de demande d’agrément et l’instruction

qui exercent sur tout le territoire, permettent aux populations les plus isolées d’avoir accès à des soins réguliers – notamment aux patients diabétiques, aux patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaires et aux patients âgés souffrant de troubles cognitifs et d’autres pathologies. Leur rôle est essentiel. Ils collaborent avec des médecins généralistes et avec tous les acteurs des soins primaires pour prendre en charge au plus près les patients, dans le cadre d’un exercice coordonné. Cette collaboration est particulièrement importante dans notre département, qui est malheureusement devenu, au fil des années, un désert médical. Cette collaboration est importante pour plusieurs raisons : elle redonne de l’autonomie aux patients sur la prise en charge de leur santé ; elle permet aux médecins généralistes de libérer du temps de consultation ; elle diminue les coûts en matière de santé. La présence de ces infirmières et infirmiers est d’un grand soutien pour les patients et elle permet aux équipes médicales de gagner un temps précieux en cas de problème

et de la prévention. Monsieur le ministre, ma question porte sur la vaccination contre le papillomavirus des jeunes dans notre pays. Le papillomavirus est une infection responsable chaque année de 6 000 nouveaux cas de cancers et de 30 000 lésions précancéreuses du col de l’utérus. Un

Et si l’on se réfère aux résultats très décevants de la première campagne de vaccination, menée dans les collèges en septembre 2023, seuls 10 % des jeunes y avaient reçu une première injection. Il y a matière à se demander pourquoi, à l’aube de la deuxième campagne, programmée pour la rentrée 2024… Je souhaite donc savoir, monsieur le ministre, si le Gouvernement dispose enfin d’un bilan précis de cette première campagne vaccinale dans les collèges, pour identifier les freins à la vaccination et en affiner les leviers. Par ailleurs, pouvez vous m’assurer de votre détermination à conduire efficacement les campagnes à venir Enfin, dans la mesure où les taux semblent différer très sensiblement d’une région à l’autre, je souhaite comprendre les inégalités entre les territoires. La région Sud, par exemple, est identifiée comme l’une des moins bien couvertes. Pour quelles raisons ? La parole est à M. le ministre

facile d’accès et qui s’apprêtent à recevoir la seconde dose. Ensuite, nous avons informé efficacement les jeunes et leurs parents de l’importance d’être vaccinés contre toute exposition au papillomavirus. Enfin, nous constatons un véritable effet d’entraînement de cette campagne au collège sur la vaccination spontanée en ville. Au total, et pour répondre très précisément à votre question, plus de 400 000 adolescents âgés de 12 ans en 2023 ont reçu au moins une dose en ville ou au collège, soit 48 % de la classe d’âge. C’est 17 points de plus que la génération précédente – celle qui avait 12 ans en 2022. Forte de ces résultats encourageants, la campagne sera renouvelée dans les collèges dès la rentrée prochaine. Notre objectif reste le même : vacciner 80 % d’une tranche d’âge d’ici à 2030, pour éradiquer les cancers liés aux HPV. Nous avons mené une évaluation interne auprès des agences régionales de santé et allons adapter le dispositif, afin de le rendre encore plus souple et plus opérationnel. Nous allons notamment renforcer l’information et la communication à plusieurs niveaux.

pour la vaccination qui aura lieu à partir de la rentrée. En outre, à la rentrée en cinquième, un second courrier d’information sera envoyé aux parents d’élèves. Parallèlement, une large campagne de communication grand public et à destination des professionnels de santé sera déployée à la rentrée scolaire. concerne, enfin, les différences territoriales, elles ne s’expliquent que par l’adhésion au vaccin, puisque cette démarche est proposée à l’ensemble des élèves, quel que soit leur lieu d’habitation.

depuis novembre dernier, l’Ehpad Les Escales du Havre, qui est le plus grand Ehpad public de France, regroupant plusieurs établissements et plus de 600 lits, est placé sous administration provisoire. La dette de l’établissement s’élève à 12,5 millions d’euros. de santé et médico sociaux propose la suppression d’une centaine de postes sur les 566 équivalents temps plein. Cela suscite évidemment et légitimement de très grandes inquiétudes parmi les soignants, qui sont déjà soumis à une charge de travail très lourde en raison de leur sous effectif. Avec une infirmière pour 120 patients, certaines unités fonctionnent en permanence en mode dégradé, ce qui affecte la qualité des soins. L’unité qui vient d’être construite fonctionnera, elle, avec un ratio d’une aide soignante pour 24 patients. patients. Ce n’est pas tenable ! Les soignants sont épuisés physiquement et psychologiquement. Ils – le plus souvent, elles, vous le savez bien – souffrent de ne pouvoir assumer convenablement l’accompagnement dû aux résidents. À ces problèmes structurels, des dysfonctionnements et des problèmes de gestion et de management se sont ajoutés, conjugués à un manque extrême de communication en direction des agents. La restructuration en cours ne fait qu’aggraver des conditions de travail déjà difficiles, avec des horaires modifiés, des personnels en moindre effectif, notamment avec le retrait annoncé du personnel de bionettoyage. La situation est vraiment délétère ; j’y insiste. Les professionnels de santé de l’établissement subissent un très grand mal être, et je crois qu’il est urgent que des mesures concrètes soient prises pour garantir la sécurité des patients et du personnel. Monsieur le ministre, quels soutiens, quelles actions quels moyens entendez vous mobiliser à titre tout à fait exceptionnel pour cet établissement, qui traverse de très grandes difficultés ? La

Les tutelles ont été alertées sur une dégradation de sa situation financière dès le mois de septembre 2023. Dès lors, l’ARS, le conseil départemental et la ville se sont mobilisés lors de réunions hebdomadaires avec l’établissement et le groupe. L’ARS a apporté des aides exceptionnelles, de plus de 3,4 millions d’euros en 2023 et de plus de 5,5 millions d’euros en 2024. Face à cette situation et au départ de la directrice, la décision des tutelles de placer l’Ehpad sous administration provisoire a été prise, en coordination avec le président du conseil d’administration. Des engagements sont prévus.

engagée au titre de la récupération de la TVA dans le cadre du chantier de travaux. Enfin, des partenariats ont été activés avec tant les acteurs du domicile que les établissements médico sociaux. Des actions de réduction des dépenses étant également nécessaires, tous les groupes de dépenses sont analysés. En matière d’exploitation, l’objectif est d’optimiser l’organisation et le fonctionnement des fonctions supports. le personnel, l’objectif est de se rapprocher des ratios, tout en assurant la qualité et la sécurité des accompagnants. Je vous annonce que l’administration provisoire donnera lieu à une prorogation à compter du 14 mai 2024, pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois.

et de la prévention. Monsieur le ministre, la Fédération de l’hospitalisation privée et les syndicats de médecins libéraux seront en grève totale et reconductible à compter du 3 juin Vous pouvez empêcher cela ! Ils déplorent la hausse de 0,3 % des tarifs hospitaliers privés en 2024, un chiffre jugé dérisoire, voire désobligeant,

assure la moitié de la chirurgie, 33 % de l’activité hospitalière et 40 % de la chirurgie du cancer. Il participe aux urgences, intervient en aval, grâce aux collaborations public privé, appréciées sur le terrain, qui limitent l’attente et optimisent les plateaux techniques. Alors que l’hôpital public est en crise, que les déserts médicaux se multiplient, que 10 % de la dette de soins héritée de la crise sanitaire est absorbée par le rebond de l’activité privée, est il judicieux d’opposer les deux systèmes ? Alors que 50 % des cliniques privées ont enregistré un déficit en 2023, qui peut croire que l’asphyxie du privé suffira à réoxygéner le public ? Les patients en seront les premières victimes, avec plus de renoncements, d’inégalités d’accès, de réductions de services, la concentration de l’offre de soins et la financiarisation dont nous ne voulons pas. Les soignants emboîteront le pas, car, en niant les efforts de gestion, en différenciant les traitements selon les exercices professionnels, l’attractivité des métiers reculera. Monsieur le ministre, les secteurs publics et privés ne sont pas concurrents : ils sont complémentaires, et la ruine de l’un ne sauvera pas l’autre. Dans mon département des Hauts de Seine, les cliniques renforcent l’hôpital public dans les services de chirurgie pédiatrique, de cancérologie ou de recherche. Mais elles jetteront l’éponge si vous maintenez votre arbitrage. Monsieur le ministre, vous êtes pragmatique. Accepterez vous une juste convergence tarifaire pour préserver le fragile équilibre du système hospitalier français ? La

depuis plusieurs années, l’État marque son engagement financier en faveur des établissements de santé, qu’ils soient publics ou privés. L’intention n’a jamais été d’opposer les uns aux autres. Depuis 2019, les ressources versées aux cliniques privées par l’assurance maladie au titre de leur activité en médecine, chirurgie et obstétrique ont augmenté de 2,2 milliards d’euros. Depuis 2021, ce sont au total 3,5 milliards d’euros de financements publics qui ont été attribués aux cliniques privées pour accompagner leurs activités et financer une partie des revalorisations salariales de leur personnel. Pour mémoire, sous la majorité précédente, entre 2013 et 2017, les tarifs pour le secteur privé lucratif ont évolué à la baisse chaque année, et cela pendant six ans. Ce n’est pas le cas cette année,

les cliniques privées comme les établissements publics ont également bénéficié en février 2024 du dispositif de soutien exceptionnel en appui à la reprise d’activité, pour un montant global de 500 millions d’euros

publics et aux cliniques privées. L’écart entre les évolutions des tarifs hospitaliers des deux secteurs en 2024 reflète essentiellement l’impact des revalorisations salariales importantes décidées depuis l’été 2023 par le Gouvernement. notamment les personnels travaillant la nuit dans les hôpitaux publics, les gardes et astreintes ayant été sérieusement accompagnées et rehaussées en septembre dernier. Cet écart des tarifs entre public et privé s’explique également par le soutien apporté par l’État à certaines

Madame la présidente, monsieur le ministre, l’allocation de solidarité spécifique (ASS) est gérée par France Travail et financée par l’État. Elle a été instaurée en 1984 pour les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage. Au début du mois de février dernier, lors de son discours de politique générale, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé la suppression de l’ASS pour les chômeurs en fin de droits, en les redirigeant vers le revenu de solidarité active (RSA).

d’abord, il s’agit une nouvelle fois d’une décision unilatérale de l’État vis à vis des collectivités territoriales, qui n’étaient pas au courant de ce projet de transfert. Cette réforme n’a donc pas été concertée avec les collectivités concernées, ce qui ne manque pas d’interpeller sur le peu de considération que le Gouvernement porte aux départements et à la décentralisation. Ensuite, et surtout, le transfert des personnes concernées par l’ASS vers le RSA aura des conséquences sur les départements. Il est en effet estimé que 300 000 personnes bénéficient de cette allocation, pour un montant de 2,1 milliards d’euros. Il n’est donc pas raisonnable de penser que ce transfert de charges se fasse sans transfert de moyens la charge financière supplémentaire que cette décision ferait peser sur les finances départementales n’est pas supportable par les départements, qui connaissent déjà « une situation d’étranglement » de leurs finances selon les termes de l’Association des départements de France. Pour l’Aveyron, le coût de cette réforme est estimé entre 6 et 7 millions d’euros par an, sans compter les moyens humains supplémentaires qui seront nécessaires à la mise en œuvre du dispositif. Monsieur le ministre, cette annonce est elle toujours d’actualité ? Les départements seront ils consultés ? L’État s’engage t il à compenser en intégralité le transfert de charges vers les départements ? La parole

contrairement au RSA, cette prestation ne peut se cumuler avec un revenu d’activité pendant plus de trois mois. En revanche, elle peut se cumuler avec des revenus du patrimoine. Est ce logique ou équitable ? L’ASS est aujourd’hui la seule prestation de solidarité qui donne des droits à retraite. Or ses conditions d’éligibilité sont complexes, et une même personne peut, ou non, avoir droit à l’ASS et aux trimestres de retraite associés, en fonction des revenus de son conjoint. Cela n’est pas équitable et cela n’incite pas, au sein des couples, à travailler plus. Comme l’a dit le Premier ministre, nous avons une conviction : la retraite doit être le fruit du travail. Mais la suppression de l’ASS se fera progressivement et ne concernera que les personnes qui pourraient entrer dans le dispositif, et non celles qui y sont déjà. C’est donc une réforme qui ne fera pas de perdants. Personne ne verra sa situation changer brutalement. J’entends enfin l’inquiétude des départements sur la charge financière supplémentaire qui leur incomberait. D’une part, je le répète, cette suppression se fera de façon très progressive. L’impact sur les départements n’est donc pas immédiat. D’autre part, cette réforme doit être analysée de façon globale, en lien avec celle de la solidarité à la source, qui conduira à la fois à faire baisser le non recours au RSA et à lutter contre la fraude et les indus, ce qui représentera aussi des économies pour les départements. La parole est à M. Jean

Monsieur le ministre, ma question porte sur les risques d’augmentation de la surpopulation carcérale durant les jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024. En effet, comme l’a récemment documenté l’Observatoire international des prisons (OIP), tous les ingrédients semblent réunis pour faire craindre une hausse substantielle des incarcérations : multiplication des patrouilles de police dans les transports à Paris, augmentation des audiences de comparution immédiate dans toutes les villes où se tiendront des épreuves et création de nouveaux délits passibles de prison au Parlement, avec la récente proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports. Parmi les établissements qui risquent d’être particulièrement touchés figure la maison d’arrêt de Villepinte en Seine Saint Denis. La situation y est pourtant déjà dramatique. Lorsque j’ai exercé mon droit de visite le 8 avril 2024, accompagnée de la bâtonnière de Seine Saint Denis, cette prison opérait avec un taux d’occupation de 180 %.

L’administration pénitentiaire compterait également sur l’ouverture du nouveau quartier centre de détention (QCD) de Fleury Mérogis. Il semblerait qu’un partenariat avec d’autres directions interrégionales des services pénitentiaires soit enfin envisagé, pour y transférer, au besoin, une cinquantaine de personnes détenues volontaires. Monsieur le ministre, ce plan d’action répond il à des instructions nationales émises par le ministère de la justice ou à des instructions régionales émises par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris ? Le garde des sceaux pourra t il me transmettre des informations précises bimensuelles jusqu’à la mi septembre 2024 sur les flux entrants et sortants au sein du centre pénitentiaire de Villepinte ? Enfin, le Gouvernement

afin d’optimiser les taux d’occupation des établissements français et de réduire la densité carcérale. En lien avec l’ensemble des structures pénitentiaires, les dix directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP) déploient une politique volontariste d’orientation des publics condamnés vers les établissements pour peine qui répond à une stratégie nationale. À ce titre, elles mettent en œuvre les opérations de désencombrement auxquelles vous faites référence. La direction interrégionale de Paris dispose de plus de 1 500 places ouvertes en droit de tirage, lui octroyant ainsi des places au sein des centres pénitentiaires d’autres DISP. Plus qu’un partenariat, ce droit permet de remédier aux déséquilibres qui peuvent exister entre les capacités d’accueil des établissements du ressort de chaque DISP. La direction de l’administration pénitentiaire (DAP) réalise aussi des opérations de désencombrement des maisons d’arrêt suroccupées vers les maisons d’arrêt ou les établissements pour peine des DISP limitrophes, lorsque c’est envisageable.

La rénovation de l’ancien quartier pour mineurs du centre pénitentiaire de Fleury Mérogis en quartier centre de détention a permis l’ouverture de 406 places. Les personnes détenues remplissant les conditions d’affectation Les personnes détenues remplissant les conditions d’affectation sont quant à elles orientées vers des structures d’accompagnement vers la sortie (SAS), telles que les SAS d’Osny et de Meaux, qui ont été livrées l’année dernière.

Mais là où cette baisse aurait pu vous conduire à entamer une révolution pédagogique, en réduisant pour tous les niveaux le nombre d’enfants par classe, et à permettre un maximum de dédoublements et de petits groupes au collège, vous fermez des classes, encore

de moyens supplémentaires. L’an dernier, vous avez fermé brutalement 178 classes dans les écoles primaires publiques et supprimé 182 postes d’enseignants dans le second degré. Pour la rentrée 2024, vous vous obstinez. Vous annoncez la fermeture de 137 classes dans le premier degré et de 58 divisions dans les collèges publics, sans compter la baisse des dotations horaires globales (DHG), qui contraint à des choix pédagogiques à rebours de l’ambition que les enseignantes et les enseignants ont pour la réussite de leurs élèves. Les collèges et lycées publics, niveau où se creusent les inégalités avec l’enseignement privé, ont pourtant plus que jamais besoin de votre soutien. Monsieur le ministre, où vont mener ces fermetures de classes sans fin, ces saignées, année après année, ces suppressions de moyens ? Écoutez ceux qui vous alertent et annulez ces suppressions de postes. Samedi

qui renvoient à des réalités incontournables. Dans l’académie de Paris, la baisse démographique s’accélère depuis plus de dix ans et affecte tous les niveaux d’enseignement. Cette déprise démographique est un phénomène structurel qui va se poursuivre. Depuis dix ans, l’académie de Paris a perdu 30 000 élèves dans le premier degré public, soit une diminution de 22 % des effectifs. Après une baisse de 2 690 élèves à la rentrée 2023, ce sont 2 031 élèves de moins qui sont attendus à la prochaine rentrée scolaire. Pour autant, l’académie de Paris détient, avec la Corse, le meilleur taux d’encadrement de France métropolitaine, avec 6,6 postes d’enseignants pour 100 élèves en 2023, contre 5,1 en 2013. Très supérieur à la moyenne nationale de 6, de 6, ce taux ferait pâlir de jalousie bien d’autres territoires. Ce taux devrait se maintenir malgré la baisse des moyens prévue et pérenniser de bonnes conditions d’enseignement pour les élèves et les professeurs. De même, le nombre moyen d’élèves par classe reste très favorable, avec 19,9 élèves en moyenne, contre 24,6 en 2013. Dans le second degré public, à l’échelle nationale, 574 créations d’emplois permettent notamment la couverture de la démographie des académies devant connaître une évolution positive. Or, à Paris, les effectifs d’élèves ont diminué de 1 443 élèves en 2023, et une nouvelle baisse de 1 276 élèves est prévue en 2024. Le nombre moyen d’heures d’enseignement par élève de l’académie de Paris, qui mesure la palette horaire dont bénéficient effectivement tous les élèves, est le reflet quasi parfait de ce même taux d’encadrement national : 1,34, contre 1,35.

comme à la rentrée 2023, chaque établissement disposera également d’une dotation dans le cadre du pacte enseignant, qui permettra la mise en place de dispositifs d’accompagnement et de soutien au bénéfice des élèves. L’académie de Paris est pleinement mobilisée, afin que tous les élèves et l’ensemble du personnel abordent la rentrée scolaire prochaine le plus sereinement possible.

En Loire Atlantique, les maires qui m’ont interpellée sur ce sujet sont respectivement cadre bancaire, agriculteur et retraité de la fonction publique territoriale. Aucun d’entre eux n’estime être à même de juger de l’état de santé

de l’enfant. Le maire, agent de l’État, a le soin de mener une enquête visant les enfants résidant sur les territoires de la commune qui reçoivent l’instruction en famille. Cette enquête doit être réalisée dès la première année, puis tous les deux ans. Son résultat est communiqué aux Dasen et aux personnes responsables de l’enfant. La loi du 24 août 2021 a modifié l’objet de l’enquête du maire. Ainsi, depuis la rentrée scolaire 2022, il s’agit pour le maire de vérifier non pas l’état de santé des enfants, mais la réalité des motifs qui ont été avancés par les personnes responsables de l’enfant.

que soit confiée à une assistante sociale de l’éducation nationale, plutôt qu’au maire, la charge de réaliser cette enquête. Toutefois, la loi ne prévoit pas que les services académiques puissent se substituer aux services municipaux pour effectuer l’enquête. Ce rôle de substitution au préfet de département. L’enquête du maire complète le contrôle pédagogique mis en œuvre par les autorités académiques, qui porte sur la qualité de l’instruction et la vérification de l’acquisition progressive par l’enfant des compétences

avait pour objet : « Apprendre à se servir des écrans et apprendre à s’en passer », j’avais formulé de nombreuses propositions pour que l’ensemble des élèves, et plus largement des citoyens, soient des acteurs actifs de leur destin numérique. Ces préconisations sont encore d’une vive actualité, à l’heure où internet et les réseaux sociaux sont devenus un espace de non droit et de menaces

de formation en écoles supérieures du professorat et de l’éducation (Espé), afin que la littératie numérique devienne un axe structurant de la formation ». Ce besoin a été le fondement de mon amendement à la loi du 26 juillet 2019, afin que les instituts nationaux du professorat et de l’éducation (Inspé) « forment les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques et à leur usage pédagogique, ainsi qu’à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique et à la sobriété numérique ». Depuis l’adoption de cette loi, à l’occasion d’auditions préalables aux lois de finances,

autorité compétente, de veiller efficacement à son respect. Toutefois, la protection des jeunes en ligne et la question de leur exposition aux écrans ne peuvent être appréhendées qu’au prisme de la sécurité. La formation des formateurs est également une clé pour relever les défis sociaux et démocratiques

a pleinement conscience des enjeux du développement des compétences numériques. Elles constituent en effet un élément essentiel du parcours scolaire, de l’insertion professionnelle et de la vie citoyenne. Depuis mars 2022, les acteurs de l’éducation nationale ont

qui fixe les trois grands axes de ce cadre de la citoyenneté numérique. Ce document est un repère des actions du ministère et de ses déclinaisons dans les académies et les établissements. Vous évoquez le, qui concerne d’abord les plateformes grand public du numérique. Il vise en particulier les plateformes des entreprises américaines des Gafam

Face aux enjeux d’éducation au numérique et de lutte contre le cyberharcèlement et afin de lutter contre les discours de haine et les contenus illicites, nous avons lancé en novembre 2022 le déploiement de l’attestation de sensibilisation aux compétences numériques à l’aide de la plateforme Pix ailleurs, la formation des enseignants est essentielle pour atteindre les objectifs fixés. La formation au et par le numérique constitue à ce titre une dimension obligatoire de la formation initiale des professeurs. Enfin, dans le cadre de la loi pour une école de la confiance, les écoles peuvent mener des expérimentations pédagogiques de cinq ans portant sur l’organisation de la classe ou de l’école, l’utilisation des outils numériques ou encore la répartition des heures d’enseignement sur l’année scolaire. Ces expérimentations sont encadrées et font systématiquement l’objet d’un suivi d’évaluation par la recherche. Le ministère de l’éducation nationale est donc pleinement engagé pour relever les défis de la formation au et par le numérique. Une approche équilibrée, progressive et sécurisée des enjeux du numérique permettra à l’école d’éduquer les futurs citoyens de demain. La parole est

de Briec, qui a organisé le week end dernier sa trente huitième Fête des fleurs, un atelier d’horticulture remarquable. Elle souhaitait ensuite appeler votre attention sur les difficultés de financement rencontrées par les Ésat, notamment dans son département. son département. Rappelons ici toute l’importance de ces lieux d’accès au travail en France, qui proposent un accompagnement spécifique pour plus de 120 000 personnes en situation de handicap. Dans la continuité du plan de transformation de ces établissements, accueilli favorablement par les structures concernées, la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi s’est inscrite dans cette dynamique positive amorcée il y a plusieurs années. Elle comprend ainsi des mesures dont la mise en œuvre doit soutenir une évolution favorable du statut des travailleurs concernés : remboursement des frais de transport public, accès aux titres restaurant et aux chèques vacances et prise en charge de la couverture complémentaire collective. de fortes inquiétudes ont été exprimées quant aux coûts additionnels induits par ces avancées, alors que la situation financière des Ésat est complexe. Plus d’un établissement sur quatre est déjà en déficit net. en déficit net. Sans soutien supplémentaire, une détérioration de l’accompagnement adapté proposé sera à déplorer, à savoir une sélection plus forte à l’entrée des travailleurs en situation de handicap, la fermeture d’ateliers moins rentables ou un temps plus restreint accordé à la formation, volet indispensable pour une insertion progressive en milieu ordinaire de travail.

Pour cela, le Gouvernement a souhaité faire converger les droits des travailleurs en Ésat avec ceux des salariés, tout en gardant la protection, spécifique à leur statut, qui empêche leur licenciement. La loi leur octroie également des droits collectifs, comme celui de faire grève ou de se syndiquer, mais aussi individuels,

fait l’objet d’un large consensus. Cependant, la mise en place d’une complémentaire santé obligatoire, prise en charge pour moitié par l’employeur, à partir du 1 juillet 2024, représente une source d’inquiétude très forte pour le secteur. À cet effet, des travaux sont en cours pour définir le meilleur moyen d’accompagner les Ésat et leurs travailleurs dans cette transition indispensable.

souveraineté alimentaire. Madame la ministre, je souhaite évoquer ici la problématique du régime spécifique d’approvisionnement (RSA), qui correspond à la compensation des surcoûts pour l’alimentation animale liée à l’éloignement et à l’absence de cultures céréalières dans les territoires ultramarins. Sachant que le coût de l’alimentation représente les deux tiers des coûts de production des éleveurs ultramarins, ce dossier a des implications majeures en matière de pouvoir d’achat de sécurité alimentaire. En outre, il nuit à l’émergence de filières de viandes biologiques dans nos départements d’outre mer (DOM), pourtant indispensables pour répondre aux obligations fixées par les lois Égalim. Le plafond du RSA n’a pas été relevé depuis dix ans et il est saturé depuis quatre À l’heure où je vous parle, ce sont 8 millions d’euros de coût de fret qui sont indûment supportés par les éleveurs des DOM, dont 5 millions d’euros pour les seuls éleveurs de La Réunion. L’État avait pourtant pris un engagement clair vis à vis de nos éleveurs : il leur a demandé de ne pas répercuter ces 8 millions d’euros sur les consommateurs. En échange, le ministère de l’agriculture s’était engagé à prendre en charge le complément du RSA, qu’il aurait obtenu le feu vert de la Commission européenne. Les éleveurs ont respecté leur engagement malgré la flambée des coûts de production consécutive à la crise de la covid 19, l’explosion du coût du fret à la fin des confinements et l’inflation galopante post guerre en Ukraine. l’État n’a pas encore respecté le sien. Bien que la Commission ait autorisé la France à verser cette aide, le ministère s’est abrité derrière le refus des collectivités locales de cofinancer ce dispositif, alors même qu’il n’en a jamais été question, et il a laissé sans réponse les nombreux courriers et les interrogations des éleveurs réunionnais. Pourtant, le Président de la République a fait de la diversification alimentaire une priorité absolue et nous a invités collectivement, le 28 février dernier, à la mettre « au centre de notre ambition agricole

de bien vouloir excuser Marc Fesneau, dont je me ferai la porte parole. Vous m’interrogez sur le régime spécifique d’approvisionnement et l’aide au fret pour les céréales destinées à l’alimentation animale. Je voudrais tout d’abord clarifier le périmètre du feu vert que la Commission européenne aurait donné à l’État, sur la prise en charge du rehaussement du plafond du régime spécifique d’approvisionnement ci a bien confirmé en juin 2023 que le rehaussement du régime spécifique d’approvisionnement pouvait être abondé par des crédits nationaux, mais cela ne signifie pas que l’État a accepté d’en verser la totalité. En effet, dans le cadre de la préparation de la visite officielle de la Première ministre à La Réunion en mai 2023, il a été décidé, concernant le financement du RSA, que le rehaussement de son plafond pour les filières animales serait pris en charge par la collectivité territoriale. Cette volonté est bien connue : un courrier cosigné des ministres chargés de l’agriculture et des outre mer a été adressé aux collectivités territoriales en août 2023. Ce courrier mettait en avant l’effort déjà consenti par l’État avec le relèvement de 15 millions d’euros des crédits du comité interministériel des outre mer (Ciom) et demandait si la collectivité voulait contribuer au développement des filières animales de son territoire par la prise en charge de l’augmentation du plafond RSA RSA et participer à la gouvernance du dispositif. Les retours des différentes collectivités sont à ce stade encore incomplets sur les montants et les périmètres de répartition des coûts entre État, région et département. Mais le Gouvernement a confirmé, en février dernier, les termes initiaux de la négociation un abondement de l’État n’est envisageable qu’à la condition d’un cofinancement de la part des collectivités territoriales. Nous restons à la disposition des collectivités pour avancer sur la définition des montants et des périmètres de répartition des coûts entre l’État, les régions et les départements. La parole

dossier que vous connaissez bien. Vous le savez, ce sujet me tient particulièrement à cœur. De l’eau a coulé sous les ponts depuis la proposition de résolution tendant au développement de l’agrivoltaïsme en France, que j’avais déposée avec mon collègue Jean Pierre Moga il y a deux ans

pour promouvoir cette forme d’agriculture durable. Malheureusement, des obstacles persistent, notamment en raison de l’arrêté du 13 mai 2023 relatif aux conditions d’éligibilité à la PAC, qui pose des difficultés majeures, en particulier du fait de la rédaction de son article 8. Ce texte impose des critères stricts, notamment celui selon lequel 30 % d’une parcelle au maximum doivent être recouverts par des panneaux photovoltaïques, ce qui entrave la liberté des agriculteurs, lesquels cherchent parfois à équiper une plus grande surface de leurs terres. Cela n’a aucun sens d’admettre l’éligibilité à la PAC des surfaces couvertes à 28 % par des panneaux, mais pas celle des surfaces couvertes à 50 De plus, les dispositions selon lesquelles l’usage non agricole doit être limité dans le temps et intervenir après la récolte ne correspondent pas à la réalité de l’agrivoltaïsme, tel qu’il se développe en France. Il est évident que les agriculteurs ne vont pas ôter leurs panneaux avant la récolte et les réinstaller quelques semaines après. Face à cette situation ubuesque, je vous interpelle sur la possibilité de prendre un arrêté modificatif, afin d’ajuster ces critères et de mieux refléter la réalité de l’agrivoltaïsme. Les agriculteurs français réclament une meilleure compatibilité entre les aides de la PAC et ces activités non agricoles. Cette demande est, je crois, en accord avec les pratiques observées chez nos voisins. Il est crucial que nous soutenions pleinement le développement de l’agrivoltaïsme en France, non seulement pour sa contribution à la transition énergétique, mais aussi pour sa capacité à promouvoir une agriculture plus durable et résiliente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Je le rappelle, l’agrivoltaïsme, tel qu’il est défini par la loi française, vise les installations photovoltaïques sur terre agricole exploitée, dont la fonction première est d’apporter un bénéfice à l’exploitation agricole amélioration des rendements ou de la qualité agronomique, protection contre des aléas climatiques tels que la grêle, économies d’eau, amélioration du bien être animal, etc. Dans ces conditions, il n’y a pas d’opposition entre production énergétique et production agricole, cette dernière étant systématiquement privilégiée. La loi APER indique explicitement que la présence d’une installation agrivoltaïque ne fait pas obstacle à l’éligibilité du terrain agricole au versement des aides la PAC. Vous avez raison de le souligner, plusieurs évolutions réglementaires sont nécessaires, dont la modification de l’arrêté définissant les conditions d’éligibilité aux aides de la PAC. Il s’agit en particulier de ne pas soumettre les projets effectivement reconnus en agrivoltaïsme à la limite du taux de 30 % de couverture que vous rappelez. S’agissant d’agrivoltaïsme, une limite de 40 % de taux de couverture a été introduite, sur la base des éléments scientifiques actuellement disponibles. Mais je rappelle que la démonstration du bénéfice agronomique est le principal critère et peut exiger, selon les situations, de s’en tenir à des taux de couverture moindres. Pour les projets en service qui répondraient à la définition de l’agrivoltaïsme, une visite par les services de l’État devra être menée rapidement, afin de confirmer le maintien de l’activité agricole et de permettre le versement des aides de la PAC. En revanche, les installations photovoltaïques au sol sur terrain agricole, qui ne sont pas agrivoltaïques dès lors qu’elles ne permettent pas le maintien strict de l’activité agricole, continueront à être soumises au régime actuel. Vous le savez, il est désormais interdit de mettre des installations photovoltaïques au sol sur des terres agricoles exploitées.

des affaires étrangères. Madame la ministre, selon l’Unicef, la bande de Gaza est aujourd’hui l’endroit le plus dangereux au monde pour un enfant. Un enfant y est blessé ou tué toutes les dix minutes, ce qui signifie que, depuis le début de cette séance de questions, six enfants ont certainement été tués ou blessés à Gaza. présent, plus de 14 000 enfants ont été tués et deux fois plus blessés, dont des milliers qui ont été amputés, souvent sans anesthésie. Des milliers d’autres sont portés disparus et sont probablement sous les décombres. En novembre dernier, le Président de la République a déclaré : « Concernant les enfants blessés ou malades de Gaza qui ont besoin de soins urgents, la France mobilise tous les moyens à sa disposition, notamment aériens,

de Gaza n’a été accueilli par la France. Seuls quelques enfants, dont le nombre est bien inférieur à celui qui avait été évoqué dans cet engagement présidentiel, ont été accueillis en provenance du Caire, où ils étaient déjà pris en soins à l’hôpital. Aujourd’hui, une quinzaine de médecins, dont deux Français, partent à Gaza dans le cadre d’une sixième mission organisée par l’association PalMed, des organismes internationaux et toujours pas par des organismes français. Aussi, que compte faire le Gouvernement pour faciliter enfin le départ de médecins français à Gaza ?

Ces besoins sont immenses. Au delà des opérations de soutien humanitaire global, plusieurs actions spécifiquement destinées aux enfants de Gaza ont été menées. Celle à laquelle vous faites référence, qui permet la prise en charge d’enfants gravement blessés au sein de nos hôpitaux, constitue sans nul doute la plus complexe. Elle doit, je crois, faire la fierté de la France. Il est important de préciser comment s’organisent concrètement ces évacuations de la bande de Gaza, qui doivent être suivies d’un transfert médicalisé, avant de déboucher sur une prise en charge hospitalière. Il s’agit

l’accord explicite des parents ou des ayants droit des enfants concernés. Nous devons, à cet égard, être en mesure de vérifier les liens de parentalité et nous assurer que le consentement a bien été donné.

Ce chiffre, qui peut vous paraître modeste, constitue pourtant une réussite importante. S’il n’est pas plus élevé, ce n’est pas parce que nous l’avons voulu – bien au contraire –, mais parce que l’hospitalisation en Égypte, ou ailleurs dans la région, est souvent privilégiée par les parents eux mêmes, pour des raisons objectives de proximité. de proximité. Nous sommes disposés et prêts à accueillir 50 enfants, comme cela avait été annoncé. De nouvelles opérations d’évacuation sont d’ailleurs en train d’être menées, en lien avec des ONG françaises qui ont sollicité notre appui pour prendre en charge des enfants nécessitant des soins lourds. La réussite de ces opérations ne doit pas être jugée à l’aune d’un seul chiffre, mais plutôt de notre capacité à organiser une intervention depuis une zone de guerre. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour la réplique.

des Français de l’étranger. La pérennité de notre système de solidarité envers les familles françaises qui ont besoin de bourses scolaires est en danger. Nous observons que les leviers pour réaliser des économies ont tous été activés : tout d’abord, l’augmentation de 2 à 7 points de la contribution progressive de solidarité a entraîné une baisse des quotités ; ensuite, l’annulation de 11,5 millions d’euros des crédits du programme 151 ; enfin, plus récemment, la baisse de l’indice de parité de pouvoir d’achat (Ippa) dans de nombreuses circonscriptions consulaires pour la campagne 2024 2025 augmente mécaniquement le reste à charge des familles. À titre d’exemple, mais je pourrais citer bien d’autres cas, l’indice est passé de 75, en 2023, à 63 cette année à Hô Chi Minh Ville, ce qui représente une baisse de plus de 8 points de quotité, alors que le taux d’inflation a atteint 4 % dans le pays. L’opacité L’opacité de cette décision, prise par le ministère sur la base de données confidentielles fournies par une agence privée, suscite l’incompréhension des conseillers des Français de l’étranger chargés d’examiner les dossiers et empêche les parlementaires d’exercer leur mission de contrôle de l’action du Gouvernement. Elle semble davantage motivée par des raisons budgétaires que par l’évolution réelle des parités de pouvoir d’achat entre la France et les pays concernés. Ce faisant, elle va à l’encontre de l’esprit même de notre système d’aide à la scolarité, conçu pour garantir l’accès de tous les élèves français à notre enseignement, quelles que soient leurs ressources financières, et pour préserver la mixité sociale au sein de l’école républicaine. Elle est même contraire aux objectifs affichés par le Président de République lui même, qui entend toujours doubler le nombre d’élèves d’ici à 2030. Madame la ministre, quels sont les critères sur lesquels s’appuie ce nouveau mode de calcul de l’Ippa ? La parole est à Mme la ministre déléguée.

Par votre question, vous sollicitez une clarification des critères mesurant l’indice de parité de pouvoir d’achat, l’Ippa, utilisé dans le barème des bourses scolaires. Cet indice est calculé à partir de données objectives fournies annuellement pour chaque poste par l’agence Mercer Consulting. Il est constitué à hauteur de 70 % de l’indice de coût de la vie et de 30 % de l’indice de coût du logement, sur la base d’un indice 100 pour Paris. Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères calcule les Ippa par poste et les transmet à l’Agence pour l’enseignement français à à l’étranger (AEFE), qui les communique aux postes diplomatiques et consulaires et les intègre au logiciel Scola de gestion des bourses scolaires. La variation de l’Ippa a une conséquence mécanique sur la valeur des aides à la scolarité qui sont versées. En effet, le contexte inflationniste mondial a entraîné en 2023 de très fortes variations. Sur 176 pays, 52 ont connu une évolution à la hausse supérieure ou égale à 10 points. Cette variation haussière a ainsi été favorable aux familles dans l’attribution des bourses scolaires pour la campagne passée. La baisse constatée dans certains postes en 2024, principalement en Afrique et en Asie, fait suite à une actualisation de la méthode de calcul des indices de coût de la vie. Celle ci a procédé, d’une part, à une mise à jour du contenu du panier de biens et de services servant au calcul de l’indice de coût de la vie et, d’autre part, à une prise en compte des charges courantes – eau, gaz, électricité, internet plus fidèle à la réalité de la consommation des ménages au niveau local. Les Ippa connaissent ainsi régulièrement des évolutions à la hausse ou à la baisse selon les pays, qui n’ont aucun lien avec des mesures budgétaires. La plupart des pays concernés par ces baisses en 2024 retrouvent en fait un indice proche de celui de la campagne 2022 2023. Les données utilisées dans le calcul de cet indice sont acquises par le ministère dans le cadre d’un marché avec Mercer Consulting, une entreprise privée. Elles ne peuvent donc pas faire l’objet d’une communication publique, car le ministère n’en est pas propriétaire.

Les lieutenants de louveterie sont des bénévoles qui assurent des missions d’intérêt général, en l’occurrence relatives à la faune sauvage, lorsque celle ci porte atteinte aux biens ou aux personnes.

qui me permet de saluer l’ensemble des lieutenants de louveterie, ces bénévoles qui assurent des missions de service public, à la demande des préfets de département, au profit des collectivités et des agriculteurs. Ils jouent un rôle essentiel en matière de régulation des espèces sauvages, de répression du braconnage et de lien social

louvetiers sont de nouveau fortement mobilisés pour la défense des troupeaux. Ils jouent, comme vous l’avez indiqué, un rôle central dans la mise en œuvre des tirs dérogatoires dans le cadre du plan national d’actions sur le loup et les activités Dans le cadre des missions relatives au loup, le défraiement et le remboursement des frais kilométriques des louvetiers sont effectifs depuis 2011. Néanmoins, en vue du renouvellement à venir des lieutenants de louveterie et de la préparation du plan national d’actions sur le loup, le Gouvernement a conduit une mission, afin d’identifier des leviers pour améliorer leur J’ai reçu les conclusions de cette mission en mars, et je puis vous annoncer, monsieur le sénateur, que je les rendrai publiques dans les prochains jours ; bien évidemment, vous en serez destinataire. Nous pourrons ainsi réfléchir

de recentrer et d’alléger leurs missions pour adapter leurs activités aux priorités actuelles, notamment celles qui sont relatives à la gestion du loup ou du sanglier. Une réflexion est par ailleurs en cours

la fin de 2022, le Défenseur des droits faisait état d’environ 500 réclamations de la part d’usagers souhaitant solliciter le dispositif MaPrimeRénov’. L’accès à cette aide financière est totalement dématérialisé pour l’usager. Il a été constaté que, faute d’équipements informatiques et d’une connexion internet pour l’ensemble des foyers français, ce seul moyen d’accès au dispositif constitue une rupture d’égalité devant le service public. Mais les difficultés ne s’arrêtent pas là. pas là. Les usagers ne sont pas les seuls à rencontrer des difficultés avec les modalités électroniques de traitement des dossiers. En effet, comme le site internet service public.fr encourage à le faire, les usagers peuvent saisir le Défenseur des droits dans le cadre de litiges avec l’administration. Ainsi celui ci est

Lancé dans le contexte particulier de la crise de la covid 19 et du plan France Relance, ce dispositif d’aide au financement des travaux de rénovation des logements est accompagné depuis le 1 janvier 2022 par le déploiement de France Rénov’, le service public de la rénovation de l’habitat, qui permet à nos

plus de 2 700 maisons France Services implantées partout dans nos territoires. Depuis 2020 et le lancement de l’aide, le Défenseur des droits a saisi l’Anah de 1 341 dossiers,

Tous les autres dossiers signalés font l’objet d’un traitement et d’une prise de contact directe avec les usagers, afin que soit trouvée une solution adaptée à chaque situation. Les équipes de l’Anah échangent

frauduleux : des propriétaires voyous se débarrassent de leurs locataires à l’approche des jeux Olympiques, pour louer leur logement pendant cette période sur des plateformes de location touristique de type Airbnb.

Ce nombre de congés frauduleux est passé en deux ans, à Paris, de 19 % à 28 %, selon l’agence départementale d’information sur le logement (Adil) de Paris.

dans leur logement, sans en être chassés par des propriétaires désireux de faire un profit maximum pendant la période des JO

dans trois cas de figure. Premier cas : le bailleur souhaite reprendre le logement pour l’occuper à titre de résidence principale ou y loger un proche. Il doit alors justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Deuxième cas : le bailleur souhaite vendre le logement inoccupé. Dans le cas d’un logement non meublé, le locataire est prioritaire pour acquérir le logement. Le bailleur doit lui donner congé en lui indiquant le prix et les conditions de la vente ; cela constitue une offre de vente. Troisième cas de figure : le bailleur met fin au bail pour un motif légitime et sérieux non respect par le locataire de l’une de ses obligations, retard répété de paiement des loyers, défaut d’entretien du logement, trouble de voisinage. En outre, la loi prévoit la possibilité pour le locataire de saisir le juge pour contester pour contester le congé. Ce dernier peut alors, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé. Il peut notamment le déclarer non valide si la non reconduction du bail ne lui apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni par une amende pénale. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de ce préjudice. Il découle de tous ces éléments que la réglementation actuellement en vigueur sur le congé est très protectrice des locataires et présente de nombreux garde fous pour limiter les abus. Il y aura toujours des gens qui fraudent,

Je suis d’autant plus inquiet que le ministre du logement passe plus de temps à expliquer comment il veut expulser que comment il compte loger. Vous lisez ses interviews comme moi tous les jours, il nous explique comment il va faciliter les expulsions locatives. Je n’ai toujours pas compris les moyens qu’il allait mettre en œuvre pour faire en sorte qu’il soit possible de se loger dans notre pays, alors même que 330 000 personnes sont à la rue et que

chargé des transports. Monsieur le secrétaire d’État, en Sud Gironde, nombreux sont celles et ceux qui doivent se déplacer vers la métropole bordelaise pour y travailler. Ils prennent leur voiture et empruntent alors l’autoroute A62. En plus du coût de leur véhicule et de l’essence, pour un trajet de Langon à Bordeaux, ils paient 4,60 euros de péage aller retour, soit 92 euros par mois, ce qui représente plus de 1 000 euros par an et par travailleur. Cette somme est énorme et injuste

des efforts sur les abonnements et le covoiturage. Finalement, c’est le que vous privilégiez. À quelques années de la fin des contrats, il est urgent que l’État ait une politique volontariste, notamment en faveur des salariés interconnectés avec les métropoles. Monsieur le secrétaire d’État, ma question est donc la suivante êtes vous favorable à l’évolution des cahiers des charges des sociétés concessionnaires pour permettre la gratuité de ces tronçons, ou en diminuer significativement les coûts ? Dans la perspective désormais urgente de la préparation du renouvellement de ces concessions, seriez vous favorable à une réduction expérimentale des coûts pour les automobilistes qui n’ont pas d’autres choix, en particulier sur l’axe Bordeaux La Réole avec l’A62 ?

par ses usagers. En particulier, le contrat de concession d’ASF, que vous avez mentionné, repose sur un péage payé par les usagers de l’autoroute A62. Toute réduction ou suppression de ce péage conduirait, ce qui est logique, à la mise en œuvre de l’obligation contractuelle de compenser le concessionnaire des pertes de recettes induites en augmentant

S’ajouterait à cela une fragilisation du péage, qui doit être proportionnel au service rendu. Or la mise à péage de cette section a été instaurée pour financer, justement, la construction de l’autoroute.

Il n’est donc pas possible d’envisager, comme vous le souhaitez, la gratuité de l’autoroute A62 entre Langon et Bordeaux dans le contexte actuel, comme cela vous a été indiqué par le ministre des transports. Pour réduire l’impact du péage pour les usagers qui empruntent quotidiennement l’autoroute, par exemple lors des trajets domicile travail, les sociétés ont mis en place depuis des années, sur la demande du Gouvernement, des formules

Le Gouvernement partage, en revanche, votre avis sur la nécessité d’anticiper la gestion du réseau autoroutier actuellement concédé après la fin des concessions historiques entre 2031 et 2036.

comment l’État compte t il participer au financement des actions de reméandrage, de création de zones d’expansion de crues ou de gestion des embâcles ? Les syndicats peuvent agir en la matière.

de Bourgogne. Ce barrage n’a pas de fonction de prévention des inondations et n’est pas dimensionné pour atténuer significativement les effets des crues de l’Armançon. Pour la sécurité de ce barrage, et donc des habitants en aval, la réglementation impose une surveillance du niveau d’eau pendant une crue. Lorsque le niveau d’eau devient élevé, le barrage doit évacuer exactement la même quantité d’eau que celle qu’il reçoit en amont. On dit que l’ouvrage devient « transparent » à la crue.

de faire en sorte que les dégâts soient les plus limités possible. Je vous remercie encore une fois de votre soutien et de votre engagement sur le sujet.

Afin de compenser les effets de la RLS depuis 2018, la construction de logements neufs a chuté de près de 100 unités par an, pour atteindre seulement 50 logements en 2023. Les réhabilitations ont décru de 20 %, passant de 900 à 750 logements, malgré les enjeux que traduit la loi Climat et Résilience. Les montants consacrés aux gros travaux d’entretien ont baissé de 2 millions d’euros. Pour leur part, de nombreux locataires sont confrontés à l’explosion des coûts lors de la régularisation des charges. Pour les 2 400 locataires de Val Touraine Habitat alimentés en chauffage collectif au gaz naturel, la facture annuelle augmente de 500 euros, voire jusqu’à 1 000 euros. L’augmentation du prix du gaz explique cette hausse, puisque le prix du mégawattheure est passé de 20,85 euros en 2022 à 141 euros en 2023. Cette situation n’est tenable ni pour le bailleur ni pour le locataire. D’ailleurs, les impayés de loyer sont passés en quatre ans de 5 % à 9 % du chiffre d’affaires de l’office. Dans ces conditions, la priorité n’est pas, monsieur le secrétaire d’État, de faire sortir du parc social les 3 % des locataires de Val Touraine Habitat, qui paient un surloyer de solidarité et qui contribuent ainsi au maintien d’une mixité sociale positive ; l’urgence est de mettre en place un tarif social de l’énergie, seule réponse adaptée à une situation qui frappe les plus modestes.

loyer modéré. Face à une crise exceptionnelle, causée notamment par la guerre en Ukraine, le Gouvernement continue d’être pleinement mobilisé pour protéger les citoyens français. Je tiens à rappeler que nous avons pris des mesures inédites pour protéger les industriels ou les particuliers. Ainsi, les ménages modestes résidant en habitat collectif ont pu profiter non seulement d’un bouclier tarifaire « individuel », qui a limité les hausses de prix du gaz et de l’électricité pour tous les contrats individuels, y compris ceux des ménages en habitat collectif, mais d’un bouclier tarifaire « collectif », qui apporte aux ménages en habitat collectif, lorsque l’électricité ou le gaz ne sont pas payés directement par eux, mais par leur copropriété ou leur bailleur, une aide équivalente à celle résultant du bouclier tarifaire des particuliers. Ces boucliers ont permis d’éviter un doublement de la facture énergétique des ménages. Les tarifs sociaux de l’énergie ont été remplacés par le chèque énergie en 2018. Ce dispositif a trois effets. Premièrement, il fait bénéficier les ménages en situation de précarité de la même aide, quelle que soit leur énergie de chauffage – électricité, gaz, fioul domestique, réseau de chaleur, bois…

Le dispositif du chèque énergie a d’ailleurs été mobilisé rapidement dans le cadre de la crise énergétique, avec l’envoi de chèques énergie exceptionnels en 2021 et en 2022 pour aider les ménages les plus modestes à payer leurs factures d’énergie. Enfin, pour la campagne 2024, le Gouvernement travaille à ce que le chèque énergie puisse être utilisé pour payer les charges locatives incluant des frais d’énergie dans le parc

introduite par amendement, sans concertation ou étude d’impact. Grâce au Sénat, ce transfert a été repoussé de 2020 au 1 janvier 2026. Depuis 2015, nous ne cessons de relancer ce sujet, avec toujours en toile de fond le souhait de plus de souplesse pour les collectivités locales. En mars 2023 a été adoptée au Sénat une proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée de ces compétences. Ce texte n’a pas été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Quelques jours plus tard, lors de la présentation du plan Eau, le Président de la République admettait sur ce sujet que « parfois, l’intercommunalité est le bon choix,

Lors des questions d’actualité du 11 avril dernier, le ministre Christophe Béchu a confirmé cet assouplissement. Un dispositif différent devrait être voté par le Parlement avant la fin de l’année et, selon ses propres mots, Sénat avant l’été. Un mois plus tard, pouvez vous nous préciser le contenu de ce projet de loi et son calendrier ? En Vendée, un collectif de maires s’est constitué sur l’initiative de Frédéric Rager, maire de Maché, et Philippe Briaud, maire de Bellevigny, dans la communauté de communes Vie et Boulogne

intracommunautaires de gestion de l’eau. L’examen du texte n’ayant pu aller à son terme, malgré un nombre très limité d’amendements, ces évolutions n’ont pas été adoptées. Néanmoins, la possibilité pour les départements de devenir membre des syndicats est inscrite dans le projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture. L’eau est une question centrale pour la souveraineté agricole de notre pays. Le Gouvernement demeure donc ouvert à la discussion, qu’il poursuit avec les parlementaires, avec vous et avec les maires de Vendée que vous avez cités, afin de permettre aux dernières collectivités qui n’ont pas encore transféré la compétence « eau et assainissement » de le faire dans de bonnes conditions.

Cette année encore, la dotation est en baisse. Il est à craindre que cela n’ait des répercussions sur les salariés, qui ne pourront plus être formés – préalable pourtant indispensable à la bonne mise en œuvre de leurs missions. Selon les dispositions réglementaires du code du travail, le plan de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés est financé par les contributions légales des entreprises, déduction faite de la part revenant aux demandeurs d’emploi. Toutefois, force est de constater un désengagement progressif de l’État au financement de la formation des salariés, au profit des demandeurs d’emploi. Les nouveaux critères de répartition des financements attribués par France Compétences posent un problème majeur pour l’avenir et pour les salariés, qui ne pourront plus bénéficier d’un parcours de développement de compétences. De plus, les structures de la branche cynégétique, essentielles au maintien et à la reconstitution de la biodiversité dans les territoires, subissent une diminution structurelle de leurs ressources financières. ressources financières. Dans quelle mesure le système de répartition des dotations de France Compétences peut il être revu afin de réattribuer la collecte des contributions légales versées par les entreprises de moins de cinquante salariés à la formation de ces derniers ?

les fédérations de chasse regroupent 1 500 collaborateurs, qui œuvrent quotidiennement dans les territoires pour encadrer et contrôler les activités liées à la chasse, surveiller et acquérir des connaissances sur la biodiversité, comme vous l’avez évoqué, et éduquer au développement durable.

Comme vous le savez, chaque branche adhérente à l’opérateur de compétences des entreprises de proximité (Opco EP) a été concernée par la modification du texte relatif à la prise en compte des salariés dans la répartition des enveloppes entre Opco, qui apprécie désormais les effectifs des branches à partir de la notion d’équivalent

EP a dû subir une baisse de 30 %. Je tiens à souligner que le Gouvernement a accompagné l’Opco pour faire face à cette situation de mise en conformité des textes en neutralisant un reversement, qui aurait dû être effectué en 2023 au titre des disponibilités excédentaires. Par ailleurs, des réunions techniques entre les équipes de l’Opco EP et de France Compétences – le répartiteur des dotations entre Opco pour le PDC – ont permis d’expliquer et de faire accepter cette méthode de calcul.

pour la prise en charge des formations en alternance dans des proportions plus importantes que pour le plan de développement des compétences. En effet, en 2023, l’Opco EP a réalisé 638 000 euros de dépenses pour les formations en alternance, contre 180 000 euros pour les formations au titre

qu’il était nécessaire de connecter la métropole lilloise et le bassin minier. Il a alors pris cet engagement : « Nous avons su nous engager pour le Grand Paris et le Grand Marseille dans des proportions massives, nous nous engagerons pour le Grand Lille, dans les mêmes proportions dès que les élus du territoire auront finalisé leur projet. » Le 13 décembre 2022, j’ai interpellé le Gouvernement sur la réalisation du réseau express Hauts de France et, une fois encore, j’ai reçu, ici même, toutes

dans la parole présidentielle. Il ne m’appartient pas de juger du mépris, de la désinvolture et du ton que le ministre a employé pour évoquer cette question essentielle pour le développement de notre territoire, mais les présidents des trois agglomérations concernées – Sylvain Robert, pour la

Au delà des démarches déjà engagées, la réalisation ou non du projet conduira à l’essor ou à la thrombose d’un territoire dont les réseaux routiers et ferrés sont saturés, le passage ou non à une économie décarbonée au pays du charbon, la volonté ou non de l’État et de ses serviteurs de respecter les élus locaux et leur engagement pour les territoires. Monsieur le secrétaire d’État, l’expression du ministre des transports est elle personnelle ou rompt elle la promesse présidentielle ?

un RER dans cette magnifique région est maintenue. Nous allons continuer de travailler avec vous pour mettre en œuvre ce projet. Ce qu’a dit Patrice Vergriete dans son échange avec les lecteurs de, c’est qu’il

De ce point de vue, la métropole de Lille et le bassin minier sont ils la bonne maille ou faut il raisonner plus largement à l’échelle de la région métropolitaine, qui inclut d’autres intercommunalités ? C’est une question que se posent d’ailleurs

évolue. Patrice Vergriete a présenté, le 23 avril dernier, le calendrier et la méthode de labellisation des services express régionaux métropolitains (Serm), en mettant l’accent sur leur périmètre et leur gouvernance. C’est dans ce cadre que les élus locaux auront à préciser les contours du projet des Hauts de France. Je n’ai aucun doute sur le fait que vous y serez Pour sa part, le Gouvernement réaffirme clairement sa volonté d’accompagner les collectivités dans leurs projets et soutient dès à présent les études et les premiers travaux, à hauteur de plus de 800 millions d’euros dans les volets « mobilités » des contrats de plan État région 2023 2027.

Il fallait évidemment bannir ce genre d’activité, particulièrement dommageable à l’environnement et contraire à la conception que nos concitoyens se font de la protection de celui ci. La loi Climat et Résilience a donc logiquement renforcé ces interdictions en prohibant les vols de transport de passagers à des fins de loisirs.

Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l’un des massifs déterminés par la loi. La liste des communes classées totalement ou partiellement en zone de montagne est ainsi fixée par plusieurs arrêtés interministériels pris entre 1974 et 1985.

de loisirs. L’édiction d’une définition différente des « zones de montagne » pour les aéronefs à moteur emporterait des conséquences sur l’ensemble des législations auxquelles la loi Montagne renvoie. Dans le souci d’assurer la clarté de la règle de droit, cela n’apparaît pas opportun.

L’interdiction de décoller et d’atterrir s’applique néanmoins si la finalité de l’embarquement ou du débarquement des passagers a un caractère récréatif ou sportif. Tel est le cas, par exemple, des activités sportives en montagne ou du transport à destination ou en provenance d’un restaurant d’altitude ou d’une résidence de villégiature

prochain, nous pourrons les interdire lors de l’examen, au Sénat, d’une proposition de loi écologiste déjà adoptée par l’Assemblée nationale. D’ici là, je souhaite interroger le Gouvernement au sujet de la pollution de l’Île de France à ces substances. Le 20 novembre 2023, l’agence régionale de santé (ARS) publiait les conclusions d’une étude menée dans vingt cinq poulaillers domestiques, à la suite des alertes lancées par le collectif 3R. Elle confirmait une contamination ubiquitaire en polluants organiques persistants (POP) et en PFAS et recommandait d’éviter la consommation d’œufs de poule issus d’élevages domestiques parisiens.

étendue à tous les territoires situés à proximité d’usines similaires, c’est à dire à une grande part du territoire national. Quels moyens le Gouvernement met il en œuvre pour expertiser la situation en Île de France, qui revêt un intérêt national ? Enfin, la presse s’est fait l’écho de défauts du contrôle des rejets de dioxines par l’incinérateur d’Ivry Paris XIII, en indiquant que des centaines d’heures d’opérations de l’usine n’auraient pas été contrôlées.

polluants organiques. L’ARS n’a cependant pas mesuré de concentrations plus importantes à proximité d’incinérateurs. Elle indique que cette contamination est probablement due à de multiples sources, comme la circulation routière ou ou les brûlages de déchets à l’air libre. Ainsi que vous le savez, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, accorde une importance particulière à ce que les incinérateurs remplissent leurs fonctions de traitement de déchets sans induire de risque sanitaire ou

le ministère a diligenté en 2024 une action de contrôle spéciale de l’inspection des installations classées sur certains incinérateurs. Plus généralement, les grands incinérateurs,

ont été respectées. Les durées d’indisponibilité de la surveillance mentionnées par les associations sont surestimées, car elles comprennent des périodes pendant lesquelles l’incinérateur était à l’arrêt, en maintenance ou en phase de démarrage sans qu’aucun déchet soit Sur le sujet plus particulier des PFAS, je souhaite rappeler que le Gouvernement est fortement mobilisé pour répondre aux enjeux environnementaux et sanitaires liés à ces substances. Il a publié le 5 avril 2024 un plan d’action interministériel sur les PFAS, qui inclut notamment l’obligation de mesurer ces substances dans les émissions des incinérateurs

Cette situation est injuste : les droits de pêche historiques, issus d’une politique de surpêche, constituent le principal critère retenu pour l’attribution des quotas, tandis environnementaux et sociaux sont à peine utilisés, au mépris de l’article 17 du règlement européen relatif à la politique commune de la pêche. Il en résulte une marginalisation systématique des pêcheurs artisans défendant de meilleures pratiques de pêche. Ce système récompense ceux qui ont la plus grande part de responsabilité dans l’effondrement des populations de poissons. Donner quelques miettes aux pêcheurs artisans et concéder l’écrasante majorité des droits de pêche aux industriels, c’est acter la mort de la petite pêche. Monsieur le secrétaire d’État, que faites vous pour protéger les ligneurs de lieu jaune ou les pêcheurs artisans de thon rouge ? Où en est l’application de l’article 17 de la politique commune ? Il y va de l’avenir des pêcheurs aux méthodes les plus responsables : ne les laissez pas couler ! La parole est

Face à cette situation, le Gouvernement a demandé aux organisations de producteurs d’effectuer un transfert de quotas au profit des navires non adhérents pour permettre à ces derniers de poursuivre leurs activités. Ce transfert entre professionnels a permis la réouverture de la pêche au lieu jaune pour les navires n’appartenant Ceux ci sont donc assurés de pouvoir pêcher pendant la période de pêche de juin et juillet : voilà une réponse concrète pour les pêcheurs artisans. Pour autant, le sujet est bien celui de la règle de répartition des quotas. Mon ministère a engagé depuis deux ans un travail de fond sur les critères d’attribution de la réserve nationale d’antériorités, constituée par les droits récupérés lors de changements d’armateurs ou de destructions de navires. Cette réserve a été alimentée à la suite de la mise en place du plan individuel d’accompagnement lié au Brexit,

La première fraction de la DSR est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton, aux communes sièges des bureaux centralisateurs ainsi qu’aux communes chefs lieux de canton au 1 janvier 2014. Cependant, l’article L. 2334 21 du même code précise que, lorsqu’une commune chef lieu de canton au 1 janvier 2014 a aujourd’hui dépassé le seuil de 10 000 habitants, les communes situées dans son unité urbaine ne peuvent plus être éligibles à la DSR,

En 2024, Groisy perdra ainsi 130 000 euros, soit près de 5 % de son budget de fonctionnement. Cette situation pénalise lourdement les communes rurales situées dans l’unité urbaine d’un chef lieu de canton ayant dépassé le seuil de 10 000 habitants. Ces communes, qui font face à des charges spécifiques liées à leur situation géographique et à leur faible densité de population, se voient privées d’une ressource financière essentielle à leur fonctionnement.

bourg centre, est destinée, par des attributions importantes, à soutenir de manière ciblée les communes supportant des charges de centralité en milieu rural. Les critères d’exclusion appliqués à cette dotation visent à prioriser les communes exerçant ce type de fonction de centralité. cas des communes de plus de 10 000 habitants chefs lieux de canton, qui assument davantage que les autres communes dudit canton les fonctions liées au maintien de services publics en milieu rural au delà de leur territoire. Venant d’un territoire rural – les Côtes d’Armor –, je sais parfaitement de quoi il retourne. C’est pour cette raison que, lorsqu’un chef lieu de canton compte plus de 10 000 habitants, les autres communes du canton ne peuvent être éligibles à la fraction bourg centre de la dotation de solidarité rurale. La création de communes nouvelles a pour objectif de créer des pôles d’attractivité dynamiques à l’échelon local, notamment en mutualisant et en centralisant les services de proximité. De ce fait, il est cohérent que le dépassement du seuil de population par la commune nouvelle chef lieu résultant d’une fusion entraîne l’inéligibilité des autres communes du canton. Par ailleurs, madame la sénatrice, je vous rappelle qu’un nouveau mécanisme en faveur des communes nouvelles a été mis en place à compter de 2023. Il permet à toutes les communes nouvelles de plus de 10 000 habitants, qui seraient considérées comme rurales au sens de la grille de densité de l’Insee, d’être potentiellement éligibles aux trois fractions de la DSR. Pour autant,

encore, c’est tant mieux, mais un certain nombre de mairies sont confrontées à des difficultés pour actualiser leurs listes d’émargement. Je m’explique : la mairie a la main sur le répertoire électoral unique

la mise en service de la téléprocédure Maprocuration en avril 2021 a permis de simplifier la procédure d’établissement des procurations de vote et d’engager sa dématérialisation. Grâce à l’interconnexion de la téléprocédure au répertoire électoral unique depuis le 1 janvier 2022, les procurations établies en ligne sont désormais automatiquement contrôlées et transmises aux communes. La gestion centralisée et informatisée des procurations dans le REU allège ainsi considérablement la charge des communes en la matière, puisque l’intervention de la mairie pour vérifier l’inscription des électeurs sur la liste électorale concernée n’est plus nécessaire, les procurations étant automatiquement inscrites sur la liste d’émargement éditée éditée à partir du REU. Dès lors qu’aucune disposition du code électoral n’impose aux électeurs de date limite pour établir une procuration à l’occasion d’un scrutin donné, il est en théorie possible d’établir une procuration jusqu’au jour des élections. En effet, cela peut impliquer de mobiliser les communes afin de vérifier la validité des procurations établies tardivement et n’apparaissant pas sur les listes d’émargement. Comme vous le soulignez, la téléprocédure Maprocuration constitue une évolution majeure en faveur de l’accès au vote, plébiscitée par les électeurs. Le droit de vote constitue un droit essentiel de nos concitoyens, qui souhaitent disposer de davantage de souplesse dans l’établissement d’une procuration.

Dès lors, le Gouvernement n’envisage pas d’imposer une date limite pour l’établissement des procurations. Cependant, des modalités pratiques d’accompagnement des communes dans la prise en compte des procurations tardives seront mises en place pour les élections européennes du 9 juin prochain, au travers d’une permanence assurée par un agent de préfecture le jour du scrutin.

La probabilité d’un recul du soutien américain dans les années à venir « sape la sécurité de tous », de l’avis même du secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg. Les leaders européens tentent quant à eux de durcir le ton face à Moscou, en insistant sur la nécessité non seulement d’aider davantage l’Ukraine, mais aussi d’augmenter leurs propres capacités de défense, car un recul du soutien américain serait dramatique. En 2023, le budget de la défense américaine représentait 67 % de l’ensemble des dépenses militaires de l’Otan. Ce pourcentage montre à quel point nous dépendons des États Unis. Parallèlement à nos propres doutes, l’Ukraine continue à subir les assauts militaires russes. Pour le seul mois de mars, elle a été frappée par plus de quatre vingt quinze missiles balistiques, et les appels au secours des dirigeants ukrainiens sur la pénurie de munitions se font de plus en plus pressants. De plus, l’Union européenne montre des difficultés à s’accorder sur sa politique de défense, ne serait ce qu’en mer Rouge, où les attaques contre des navires marchands européens se multiplient depuis décembre. Madame la secrétaire d’État, ma question résonne avec le calendrier électoral : quelle défense européenne voulons nous ? Quel mode de gouvernance efficace voulons nous dans ce monde instable, où la résurgence de nombreuses menaces inquiète les populations de notre continent européen ?

équipées, interopérables et immédiatement déployables, en faisant en sorte que 2 % de notre PIB soit réellement utiles militairement. De plus, en matière de préparation à la mission de défense collective, l’Otan offre un processus de planification capacitaire membres sur le long terme. Les accords dits Berlin plus prévoient des capacités de commandement et de contrôle utilisables dans le cadre d’un mandat de l’Union européenne ainsi qu’une standardisation et un processus de certification des forces à l’échelle du niveau d’ambition d’un conflit majeur sur le continent européen. Par ailleurs, l’Union européenne travaille efficacement dans des domaines connexes. Par exemple, dans le cas de l’Ukraine, nous assurons des formations militaires ou la construction de coalitions capacitaires et industrielles, dans l’esprit de l’initiative lancée par le Président de la République.

Enfin, la France mène une politique de réarmement qui contribue indéniablement à la défense de l’Union européenne. Sous l’impulsion du Président de la République, au terme de deux lois de programmation militaire, la France aura doublé son budget de défense entre 2017 et 2030. Pour la période 2024 2030, cela représente des augmentations cumulatives d’au moins 3,2 milliards d’euros par an. La France consacre 29 % de ses dépenses de défense à l’investissement, à la fois dans ses moyens conventionnels et dans la modernisation de sa dissuasion nucléaire. Nous devons continuer à avancer en Européens. La parole

indiquer, dans un rapport, l’état de partage des sites mobiles. De plus, avant toute implantation d’antenne, un temps de dialogue le dépôt des dossiers d’informations au maire est requis. En principe, rien n’est fait à l’encontre des décisions du maire et sans concertation locale.

les parlementaires de tous bords politiques à trouver de nouvelles recettes fiscales. Pourtant, madame la secrétaire d’État, malgré l’implication concrète des parlementaires, nous avons le sentiment que votre gouvernement n’écoute pas les propositions qui lui sont faites.

M. Jean Paul Mattei, président du groupe centriste à l’Assemblée nationale, tout comme de nombreuses figures du groupe Renaissance, fait valoir qu’il est possible de prendre des mesures de justice sociale sans pour autant briser la croissance. Madame la secrétaire d’État, pour éviter que le pays ne bascule dans le camp de l’extrême droite, il est nécessaire de rétablir de la justice sociale,

Il y a urgence à agir, d’autant que – nous venons de l’apprendre – la Commission européenne devrait placer la France sous procédure concernant ses déficits excessifs. Ma question est donc simple : envisagez vous de modifier le niveau de taxation des Français les plus aisés afin de rétablir une certaine équité et de sortir notre pays de l’impasse budgétaire dans laquelle il se trouve ?

atteint ses objectifs : elle porte aujourd’hui ses fruits. Vous le savez, pour la cinquième année consécutive, la France est en 2023 le pays d’Europe qui a attiré le plus grand nombre d’investissements étrangers. Depuis 2017, nous avons réussi à créer 2 millions d’emplois, le secteur industriel. La réindustrialisation du pays est bien en marche, 200 nouvelles usines ayant été ouvertes en France en sept ans. Ces résultats, monsieur le sénateur, nous les avons obtenus en baissant les impôts, sur les ménages comme sur les entreprises, à hauteur de 60 milliards d’euros. en effet convaincus d’une chose : c’est par la croissance et par l’emploi que nous pourrons financer nos priorités. Ces emplois, ces usines et toute l’attractivité ainsi créée sont les recettes fiscales d’aujourd’hui. Nous souhaitons poursuivre cette politique. Mais nous savons aussi nous adapter. Ainsi, c’est pour répondre aux situations exceptionnelles liées aux crises récentes que le Premier ministre a confié à plusieurs députés de la majorité le soin de faire des propositions de mesures fiscales spécifiques – nous attendons le fruit de leurs travaux. Nous avons également agi à l’échelon européen : en témoignent la mise en œuvre d’une taxation des géants du numérique

les entreprises du secteur du tourisme de plein air ont construit des zones de baignade dans le but d’offrir aux vacanciers, de plus en plus exigeants en la matière, des équipements d’excellence. de leur rendre hommage, tant l’enjeu est essentiel pour l’attractivité de nos territoires : l’hôtellerie de plein air et les PRL représentent en France plus de 30 % de l’offre de vacances. Mais

Le Conseil d’État a précisé, le 25 juillet 2007, que l’obligation de surveillance doit être respectée dès lors que le bassin n’est pas réservé à une clientèle propre. Or, dans le cadre d’une piscine réservée à la clientèle d’un PRL, la piscine est qualifiée de « privée à

est à Mme la secrétaire d’État. Madame la sénatrice Delattre, la réglementation relative aux piscines privées à usage collectif concerne les piscines dont l’accès est réservé à un public restreint identifié du fait d’une autre prestation prestation de service principale, sans lien direct avec la pratique d’une activité physique et sportive. Il s’agit notamment des piscines d’hôtel, de restaurant, de camping et de village de vacances, dotées d’une clientèle propre et dont l’ouverture n’est pas Cependant, afin de garantir au mieux la sécurité et la qualité de la prestation offerte, une surveillance peut y être mise en place. Le cas échéant, l’exploitant devra mettre à disposition du personnel qualifié ainsi mobilisé l’ensemble des moyens nécessaires au secours. Le Conseil d’État, dans un avis rendu le 26 janvier 1993,

une surveillance constante par du personnel qualifié, conformément à la législation en vigueur. Ces établissements sont par ailleurs soumis à certaines obligations administratives : l’exploitant doit avertir ses usagers de l’éventuelle absence de surveillance de la baignade, de la responsabilité des utilisateurs, des heures d’ouverture et du règlement intérieur du bassin ; il doit souscrire un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle de ses préposés et celle du public ; il doit réaliser un affichage, entre autres, du règlement intérieur, du plan de sécurité, des profondeurs, du mode d’emploi des équipements et du contrat d’assurance en responsabilité civile. l’un des quatre dispositifs de sécurité normalisés – barrière de protection, couverture, abri ou alarme – doit être mis en place. Autrement dit, rien n’interdit aujourd’hui de mutualiser l’accès à une piscine, dès lors que les personnes pouvant y accéder sont clairement identifiées. L’obligation de surveillance trouvera

comptable censé évaluer la qualité de la gestion comptable de la commune. Tout en précisant que ce document ne vaut pas jugement de la gestion de la collectivité, la DGFiP délivre néanmoins une note d’identifier les marges de progression, les points forts et les points faibles de la tenue des comptes locaux. Vous comprendrez, je l’imagine, le caractère irritant de ce mode d’évaluation

N’est ce pas aux élus locaux d’évaluer l’efficacité des politiques publiques et de fixer les orientations aux fonctionnaires, et non l’inverse ? C’est normalement le service de gestion comptable qui est responsable de la qualité comptable, puisqu’il tient, avec l’élu, le compte financier unique. Or l’avis critique du conseiller aux décideurs locaux sur le travail de son collègue comptable remet en cause la compétence exclusive de ce dernier en imposant une orientation à suivre. Un tel avis est clairement perçu comme une forme d’ingérence des services de l’État qui contrevient,

produit depuis 2020 par la direction générale des finances publiques pour remplacer l’ancien indicateur de qualité des comptes locaux. Cet indicateur rénové vise à mesurer les conditions d’application de la réglementation budgétaire et comptable. Il est fondé sur les résultats,

aisément évocatrice. Monsieur le sénateur, cet indicateur ne vise nullement à se prononcer sur la qualité de la gestion d’une collectivité, sur la qualité de son financement ou sur sa solidité financière. il ne prend en compte ni l’environnement de maîtrise des risques ni les conditions de déploiement des dispositifs de contrôle interne et comptable des collectivités locales. La visibilité offerte à cet indicateur, souhaitée par le Comité national de fiabilité fiabilité des comptes publics locaux, représente un levier important de l’amélioration de la qualité comptable pour toutes les collectivités territoriales. L’IPC doit donc être appréhendé comme un outil partagé entre l’ordonnateur et le comptable, permettant de cibler des actions à en vue d’améliorer la qualité du processus comptable. Il offre un éclairage sur la comptabilité de chaque collectivité et de chaque budget, mettant en évidence un certain nombre de points forts et de points faibles ; ainsi permet il d’identifier les marges de progression et de suivre les améliorations apportées. Il ne constitue pas un label de qualité des comptes ni un critère exclusif d’appréciation de leur fiabilité, mais doit être intégré avec d’autres données dans une démarche progressive et plus globale d’amélioration de la qualité des comptes. Les comptables publics ou les conseillers aux décideurs locaux peuvent également proposer aux ordonnateurs la réalisation d’une synthèse de la qualité des comptes de l’exercice clos, dont les résultats sont partagés avec l’ordonnateur et présentés aux élus à l’occasion de l’adoption

TVA. La fabrication et la vente de biens neufs par les opérateurs économiques sont normalement soumises à la TVA, sans que la nature des matières premières ou le régime fiscal qui leur a été appliqué dans le cadre d’un cycle de consommation finale antérieur

été acquis auprès de particuliers et à la condition que les modifications apportées au bien revendu se limitent à une remise en état et non à sa transformation en un objet nouveau. Par ailleurs, l’application de taux réduits de TVA est strictement encadrée par la directive précitée, les États membres de l’Union européenne ne pouvant appliquer pareils taux qu’à certaines catégories de biens certaines catégories de biens ou de services. Or il n’existe aucune disposition autorisant un État membre de l’Union européenne à appliquer un tel taux réduit aux ventes de biens résultant d’un circuit de recyclage. Aussi la vente d’accessoires vestimentaires neufs ou recyclés est elle soumise de plein droit au taux normal de Au delà de ces considérations juridiques, monsieur le sénateur, l’expérience a montré que les baisses de taux de TVA sur certains produits ont un coût significatif pour les finances publiques sans pour autant, malheureusement, constituer des leviers efficaces : elles donnent rarement lieu à une baisse des prix au profit des consommateurs.

pilotés par les préfets et par le ministère des transports sur chaque site accueillant des épreuves. Le préfet de police a d’ailleurs pris la parole, le 25 avril, pour détailler les mesures de sécurisation qui seront déployées en amont de la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques.

Les panneaux solaires chinois, qui sont en moyenne quatre fois moins chers que les produits français, envahissent par conséquent le marché. Les prix des panneaux solaires vendus en Europe ont dû diminuer de 25 % depuis janvier 2023, menaçant de nombreuses entreprises françaises. Cette stratégie chinoise est totalement contraire aux règles édictées par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ; elle met en péril les efforts que déploient l’Union européenne et la France dans leur volonté d’autonomie énergétique et de réindustrialisation, que nous sommes nombreux à partager. Les dispositifs réglementaires qui permettraient de restaurer une compétition loyale entre les différents acteurs industriels tardent malheureusement à être mis en œuvre. Ils n’auront pas d’effet dans un délai compatible avec les enjeux qu’ont à relever les entreprises françaises, lesquelles réclament une action politique immédiate.

de la stratégie énergétique et industrielle du Gouvernement. Il y a là un impératif si l’on veut sortir des énergies fossiles sans remplacer une dépendance par une autre : produire, pour notre souveraineté, les équipements de l’éolien, du photovoltaïque, des pompes à chaleur, ce qui veut dire notamment Le photovoltaïque a une place importante au sein de la réindustrialisation verte que nous souhaitons. Nous visons en la matière la multiplication par cinq, dans les dix ans à venir, des capacités installées, ce qui représente 20 milliards d’euros d’investissements partout sur le territoire. Pour répondre à cette demande, deux acteurs historiques continuent de produire des panneaux et deux sont en développement – elles produiront dès 2026 leurs premiers panneaux et couvriront, nous l’espérons, nos besoins nationaux. L’enjeu est de préserver la viabilité économique de ces projets face à la chute des prix des panneaux chinois enregistrée en 2023, qui s’inscrit dans une stratégie commerciale agressive plus globale de notre partenaire. cette fin, le Gouvernement déploie plusieurs actions. Premièrement, en amont, pour soutenir l’investissement, nous avons mis en place un crédit d’impôt qui couvrira jusqu’à 200 millions d’euros d’investissements par projet. Deuxièmement, en aval, pour favoriser l’installation de panneaux produits en Europe, nous faisons évoluer dès cette année les critères d’attribution des tarifs d’achat : une prime sera versée pour les panneaux les plus vertueux sur le plan environnemental. Troisièmement, nous mettrons en œuvre dès 2025 les dispositions du, le règlement pour une industrie « zéro net », que nous avons négocié à Bruxelles, en orientant les subventions publiques vers des projets projets qui concourent à la résilience de l’économie européenne. Enfin, sur l’initiative du Gouvernement, les acteurs se sont engagés dans un pacte de solidarité de filière. Les acheteurs participeront à la sécurisation des nouvelles usines par des commandes passées à l’avance et nous mettons en place l’« induscore », qui tracera le nombre d’étapes de fabrication réalisées en Europe.

Ces établissements d’accueil temporaire ou permanent agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée peuvent bénéficier d’un taux de TVA réduit de 5,5 % sur leurs travaux d’extension dès lors que ceux ci sont affectés à de l’habitation pour au moins 50 % de la superficie.

Compte tenu de la volonté unanimement exprimée de réduire les procédures administratives, ne serait il pas opportun d’alléger les démarches en imposant dès le départ une taxation au taux de 5,5 %, afin d’éviter des jeux de trésorerie synonymes de coûts, de tracasseries et de perte de temps ? de temps ? Ce taux de TVA de 5,5 % peut il s’appliquer de manière directe dans le cadre d’une « contractance » générale ? Madame la secrétaire d’État, le Gouvernement serait il prêt à prendre des dispositions destinées à simplifier ce dispositif ?

Quant aux Ehpad gérés par des personnes morales de droit privé, qu’ils soient ou non à but lucratif, ils sont assujettis à la TVA, mais bénéficient, sous certaines conditions, du taux réduit de 5,5 % pour leurs prestations d’hébergement ainsi que d’une exonération de la TVA pour la partie de leur activité correspondant aux aux soins fournis aux personnes hébergées. Lorsque ces établissements font édifier des locaux neufs ou procèdent à des extensions de locaux, ces constructions bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 % au titre de la taxation de la livraison à soi même

si le fait générateur de la taxation de la livraison à soi même intervient à la date de l’achèvement des travaux, le législateur a prévu que la liquidation de la TVA au taux réduit de 5,5 % intervienne au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette même date. En revanche, la déduction peut se faire dès le mois suivant la fin de ces travaux.

les départements où la taxe de séjour est la plus faible, ce qui risque d’avoir un impact sur le tourisme d’affaires. Cela relève du bon sens que les hébergeurs des établissements dont le territoire est limitrophe des régions périphériques de l’Île de France, comme le Centre Val de Loire ou les Hauts de France, puissent bénéficier d’une adaptation du dispositif une exonération pérenne ou tout autre levier permettant d’éviter la création

représente un faible surcoût pour les voyageurs » rapporté au coût d’une nuitée et que « peu d’effets macroéconomiques significatifs sont à attendre ». Par exemple, la taxe additionnelle de séjour sera au maximum de 9,20 pour un palace parisien, de 5 euros pour un hôtel quatre étoiles et de 3,20 euros pour un trois étoiles. Cette taxe additionnelle, dont le taux a fait l’objet d’une large concertation avec les représentants de l’hôtellerie, doit rapporter environ 200 millions d’euros par an. Cela permettra d’aligner la région capitale sur les standards d’autres capitales européennes La distorsion de concurrence que vous redoutez, par exemple entre les hébergements situés en Essonne et ceux qui se trouvent en région Centre Val de Loire, semble limitée eu égard au montant de la surtaxe par nuitée, en particulier pour la clientèle d’affaires présente dans le département de l’Essonne.

que de façon marginale. Il ne me semble pas logique que les territoires éloignés de la métropole parisienne, qui assurent par ailleurs une partie non négligeable de son financement sans bénéficier de ses retombées, subissent une double peine, puisque cette taxe additionnelle nuit aussi à leur attractivité. La parole est à M. Pierre Antoine

Alors que la prospérité bat à notre porte, nous restons, par un choix mystérieusement volontaire, en marge de cette richesse potentielle. Il est singulier, voire troublant, de constater que tandis que nos voisins se préparent à récolter les fruits d’un eldorado noir, la Guyane française ne semble pas avoir choisi cette option. N’est il pas paradoxal, madame la secrétaire d’État, que la nature ait distribué ses faveurs avec tant de générosité autour de nous et que seul notre territoire semble exempt de cette manne ? Cette situation interroge : sommes nous face à une absence réelle de ressources ou plutôt à une volonté délibérée de ne pas explorer, de ne pas chercher ? Il apparaît comme une incongruité géologique que la Guyane soit la seule terre vierge de cet or noir dans une région en pleine effervescence extractive. Ce choix – si c’en est un – de ne pas engager notre territoire dans la course à l’exploitation pétrolière mérite d’être scruté avec la plus grande attention. Il soulève une question de justice et d’équité pour les Guyanais, qui observent, impuissants, leurs voisins s’enrichir. Comment expliquer à nos concitoyens que nous restons les bras croisés alors que, potentiellement, des richesses sommeillent sous nos pieds ? En omettant volontairement de rechercher ou d’exploiter d’éventuelles ressources pétrolières en Guyane, ne sommes nous pas en train de condamner notre territoire à l’isolement économique ? Quelle ironie ce serait que de voir un jour le Guyana, enrichi par ses hydrocarbures, venir en aide à la Guyane française, oubliée de la prospérité pétrolière.

C’est pourquoi la France s’est engagée, par la loi dite Hulot de 2017, à interdire la délivrance de nouveaux permis de recherches d’hydrocarbures et à ramener à 2040 la date de fin des concessions existantes. La France a renforcé son engagement dans l’accord de Paris

que nous avons pris. L’interdiction d’exploration introduite par cette loi garde sa pertinence sur la totalité du territoire national. Par ailleurs, la politique menée par la France vise une réduction importante de la part des hydrocarbures dans notre mix énergétique d’ici à 2045. L’exploration

et à une exploitation déterminée des ressources naturelles minières de la Guyane, au service du développement économique du territoire. Le projet de loi de simplification de la vie économique comprendra d’ailleurs des dispositions de simplification de l’exploration minière sur l’ensemble du territoire national, ainsi que des dispositions spécifiques aux autorisations minières les plus utilisées en Guyane, pour faciliter l’exploitation minière dans ce territoire au sous sol très riche. La parole

directement touchés par cet arrêt brutal. Nous pourrions rester indifférents à cette situation, mais, élue du territoire, je suis évidemment en totale solidarité avec les salariés, leurs proches, les habitants

de nouveaux secteurs de la chimie, tels que le recyclage moléculaire ou le bioraffinage, avec notamment l’implantation de l’américain Eastman et du belge Futerro, qui fabriqueront le plastique des prochaines décennies, dégradables, mais aussi biosourcés.

et nous serons extrêmement vigilants quant aux projets d’investissements à venir sur ce site. Nous en